La séance est reprise. Les conclusions adoptées par la conférence des présidents réunie ce jour et complétant l'ordre du jour établi lors de la réunion de la conférence des présidents du 7 novembre 2018 sont consultables sur le site du Sénat.

n'est pas parvenue à l'adoption d'un texte commun. Je l'informe également que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 n'est pas parvenue à l'adoption d'un texte commun.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 citoyen et écologiste, sur les conditions de mise en oeuvre de l'accord économique et commercial global, ou CETA. Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents.

mon groupe a souhaité ce débat sur les conditions de la mise en oeuvre du CETA, ce traité de libre-échange conclu entre l'Union européenne et le Canada, pour une raison, somme toute, assez simple : il règne une grande opacité autour de ce traité de nouvelle génération opacité dans sa négociation, dans sa mise en oeuvre, quant à ses effets et, enfin, dans l'échéance de sa ratification. Effectivement, ce traité n'est pas un accord commercial comme un autre.

son enjeu majeur est de viser également à amoindrir toutes les entraves existantes au commerce, même lorsqu'est en jeu l'intérêt général, avec notamment nos services publics, notre santé et l'environnement. C'est ce que l'on appelle les barrières non tarifaires. Ce débat devient urgent, car de nouveaux traités sont en préparation, avec Singapour, le Mercosur, le Vietnam, l'Indonésie, ou encore le Japon- le JEFTA ; il y en a quinze sur la table. Or, pour débattre en toute connaissance de cause, nous avons besoin d'études d'impact sérieuses sur ce type de traités, dont nous ne connaissons pas encore suffisamment les effets. Je parlais d'opacité ; le CETA a été négocié à Bruxelles, au troisième sous-sol, par la Commission européenne de 2006 à 2014. Même si, depuis lors, nous avons gagné en transparence sur les mandats de négociation, avec notamment leur publication sur le site du Parlement européen, ... Tout à fait ! ... et, même si l'Union européenne a toute compétence pour ces négociations depuis le traité de Lisbonne, la question de l'association des parlements nationaux reste, selon nous, un enjeu majeur. Le CETA, signé le 30 octobre 2016, est entré en vigueur de manière provisoire le 21 septembre 2017 pour sa partie relative aux barrières tarifaires. Nous devions nous prononcer sur la question des barrières non tarifaires, car celles-ci modifient profondément les législations européenne et nationale. Or comment serait-il possible

un mieux-disant social et environnemental. Or, du côté canadien, les experts insistent sur l'absence de garanties concernant les farines animales, les antibiotiques comme activateurs de croissance, l'étiquetage des produits contenant des OGM et le type et les niveaux de pesticides autorisés.

ce n'est en rien surprenant, les hormones étant autorisées dans l'élevage au Canada ; la mise en place d'une filière sans hormones, destinée à l'export, prend du temps. Pour autant, sans hormones » ne signifie pas sans antibiotiques ni sans mauvais traitements. De plus, l'Union européenne et le Canada ne sont pas d'accord sur la reconnaissance automatique de leurs standards phytosanitaires. Enfin, les contingents canadiens atteindront leur plein potentiel en 2023, conformément à cet accord. Il s'agit d'une concurrence déloyale pour notre agriculture et de la mort, à terme, de notre agriculture paysanne.

se retrouvera pas un jour dans nos assiettes ? Les risques ne sont donc pas écartés, et nous ne pouvons pas ne pas les évoquer. Nous parlons de risques, mais le climat est le grand oublié de ce traité. Un rapport commandé par les gouvernements prévoyait une hausse des émissions de gaz à effet de serre, du fait de l'augmentation de 7 % du trafic maritime entre l'Europe et le Canada, et de la promotion des investissements dans des industries polluantes, celle du pétrole issu des sables bitumineux. Sommes-nous donc toujours coincés dans la logique « pas chez moi, mais ailleurs, pas de problème, allez-y, polluez ! » ? Nous bannissons ou nous atténuons ici des pratiques pour en les cautionnant par l'importation ! Alors que les émissions de gaz à effet de serre ont de nouveau augmenté en 2017, de 3,2 %, nous voudrions poursuivre ce mouvement destructeur ? Cela n'a absolument aucun sens. Nous n'avons pas non plus de nouvelles concernant le veto climatique annoncé voilà un an. Bref, les incohérences sont flagrantes, sans parler de l'actualité, comme le forage ou le projet Montagne d'or en Guyane.

nier aux parlementaires le droit de se prononcer sur le CETA ? Ce traité a été ratifié du côté canadien et par le Parlement européen. Chacun des États membres devait ensuite le ratifier, ce qu'ont fait la Lituanie, la Lettonie, le Danemark, la Croatie et le Portugal. En France, la ratification devait intervenir un an après la mise en oeuvre provisoire.

à nous prononcer ? Pour laisser le temps au gouvernement italien de trouver les moyens d'approuver ce traité, afin de ne pas compromettre son adoption ? En effet, rappelons-le, il suffit qu'un seul des États membres le rejette pour que cet accord tombe de lui-même. Monsieur le secrétaire d'État, une vraie question

de débat public et de réelle information des citoyens, qui doivent pouvoir décider en toute connaissance de cause. Un choix qu'il s'agirait de respecter véritablement, contrairement à ce qu'il s'est que ce soit l'un des enjeux des prochaines élections européennes, et peut-être, monsieur le secrétaire d'État, pourriez-vous l'inclure dans le clip de propagande gouvernementale que vous diffusez actuellement

qui seront au-dessus des États et donc de leurs lois, ce qui nous concerne en tant que citoyens, mais aussi en tant que législateur. Allons-nous laisser les laisser les multinationales attaquer nos États et nos lois, celles que nous votons ici pour défendre les Françaises et Français, notre agriculture, nos entreprises, notre modèle social Les Amis de la terre a récemment révélé qu'une entreprise canadienne, Vermillon, avait menacé l'État français de poursuites sur le fondement d'un autre accord de protection des investissements pour amoindrir, avec succès, la portée de la loi Hulot sur la fin de l'exploitation des hydrocarbures. Je sais que cette loi a fait débat, mais je suis certain que chacun a à coeur que la décision que nous avons adoptée ne soit pas remise en cause par le pouvoir économique, car cela signifierait la fin du pouvoir politique. La société de demain doit-elle être administrée par les entreprises GAFAM et par les multinationales ? démissionnons et déplaçons l'hémicycle dans leurs conseils d'administration, cela ira plus vite ! Nous vous proposerons, mes chers collègues, de nous opposer ensemble à cette disposition. Si vous me le permettez, madame la présidente, j'aimerais finir

tandis que le système du libre-échange est destructeur. Il dissout les anciennes nationalités et pousse à l'extrême l'antagonisme entre la bourgeoisie et le prolétariat. En un mot, le système de la liberté commerciale

vous ne m'aurez pas l'usure ; au contraire. Il y a une volonté intacte de pouvoir conduire à bien ce chantier, qui va très clairement conforter la relation entre la France et le Canada, entre l'Union européenne et le Canada.

le Canada est un partenaire important pour la défense du multilatéralisme. Voilà quelques jours, nos amis canadiens accueillaient à Ottawa une conférence sur l'avenir de l'OMC,

permet d'assurer le respect strict de nos normes. Tout produit importé au sein de l'Union européenne doit impérativement être sûr, ne présenter aucun danger pour la santé des consommateurs et respecter les normes dont nous nous sommes dotés, comme l'interdiction de produits OGM.

chaque orateur peut intervenir pour deux minutes maximum pour présenter sa question, avec une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente. Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de trente secondes supplémentaires,

de la mise en oeuvre du CETA. Si les exportations vers le Canada sont globalement en hausse, notamment le chocolat belge, le jambon italien, mais aussi les fromages, les fruits ou les produits pharmaceutiques, ce fait ne doit pas masquer des réalités plus dérangeantes, notamment pour certains produits français qui subissent des pratiques commerciales

encore que l'Ontario applique des taxes de 60 centimes de dollars canadiens par litre, tandis que les vins nord-américains ou chiliens bénéficieraient de réductions de 30 centimes par litre. Je vous invite à vérifier ces faits, qui montrent que la situation des vins et spiritueux européens au Canada s'est globalement détériorée ces derniers mois.

Connaissant les difficultés que rencontre la filière, cette situation est inacceptable. Monsieur le secrétaire d'État, fort de ces constats, comment pensez-vous protéger les intérêts des agriculteurs français ? Notre modèle familial est particulièrement respectueux de l'environnement. Envisagez-vous de faire valoir l'exception pour le secteur sensible de la viande bovine ?

Il a pour objectif de dynamiser les échanges commerciaux entre l'Union européenne et le Canada, d'accroître la croissance, de créer des emplois et de nouveaux débouchés pour les entreprises européennes et françaises. En effet, l'Union européenne et le Canada nous ont promis d'établir une communication continue et transparente. Le Canada publiera tous ses appels d'offres sur un site web consacré aux marchés publics. Ce site aidera les PME françaises, puisque l'accès à l'information est l'un des principaux obstacles auxquels elles sont confrontées pour accéder aux marchés internationaux. Vous nous avez dit voilà quelques instants, monsieur le secrétaire d'État, que les premiers résultats étaient encourageants. Le présent débat nous offre aussi et surtout l'opportunité de dresser un bilan de la façon dont l'Union européenne négocie pour nous les accords commerciaux, puisque c'est l'une de ses compétences exclusives. D'une manière générale, je pense que la Commission devrait mieux prendre en compte les spécificités des régions ultrapériphériques, comme l'a souligné un précédent orateur. Les grands accords commerciaux peuvent en effet avoir un effet désastreux sur les producteurs locaux dans nos outre-mer. Il faut y veiller, alors que nous allons signer des accords avec l'Amérique latine ou l'Australie. Il me semble également que les enjeux climatiques et de développement durable devraient davantage être inclus dans nos accords. Le commerce doit être un levier européen pour étendre ses standards de protection de l'environnement au monde entier. Enfin, il convient de s'assurer d'une meilleure réciprocité avec nos partenaires. Sans sombrer dans un protectionnisme stérile, il est fondamental que l'Europe réagisse et prenne des mesures pour faire face aux États-Unis ou à la Chine qui renforcent leurs instruments de défense commerciale ou bloquent l'accès à leurs marchés publics. L'Union européenne ne peut se permettre d'être naïve sur les enjeux commerciaux, alors qu'elle est la troisième puissance commerciale du monde. Le Canada est un pays riche en ressources naturelles et constitue un vaste marché, essentiel pour les exportations européennes. L'Europe la France en ont besoin, mais pas à n'importe quel prix. Je voudrais donc savoir, monsieur le secrétaire d'État, quelle position défendra la France pour moderniser la politique commerciale de l'Union européenne à la lumière du bilan du CETA.

les barrières non tarifaires seront levées plus facilement pour des biens qui contribuent à la lutte contre le changement climatique, à la protection de l'environnement. Nous nous inscrivons bien dans cette ambition affirmée. Quant à la réciprocité, vous parlez d'or.

dans un objectif de protection des consommateurs et de notre filière agricole. Dans le même temps, la France ouvre de plus en plus son marché à des denrées provenant de pays aux exigences différentes. À ce titre, le CETA permet au Canada

Les négociations entre l'Union européenne et le Mercosur pourraient, quant à elles, autoriser l'importation de 99 000 tonnes de viande non tracée, issue d'élevages utilisant de manière intensive les antibiotiques et les farines animales.

d'État, je m'interroge sur le manque de vision globale de la politique commerciale extérieure de la France et de l'Union européenne : le Parlement s'engage en faveur de la protection des consommateurs et de la filière agricole et, dans le même temps, le Gouvernement donne à la Commission européenne un total blanc-seing pour négocier, sans que la France soit directement impliquée, une multitude d'accords ouvrant de larges brèches dans notre système de surveillance sanitaire. Il y a un vrai déficit d'évaluation des conséquences de chaque accord sur les filières. L'effet cumulé de ces différents accords bilatéraux n'est pas non plus étudié. Monsieur le secrétaire d'État, comment assurer que nous connaissons l'impact global sur chaque filière de l'ensemble des accords et comment en évaluer les conséquences au moment où les frontières

peser dans les discussions auprès de la Commission. La question de l'impact cumulé est un combat que nous menons de longue date, de pair avec nos amis belges.

M. Guillaume Gontard. Monsieur le secrétaire d'État, le 14 février dernier, Nicolas Hulot déclarait à l'Assemblée nationale que le CETA et le Mercosur « ne sont pas en l'état climato-compatibles ». Cette lucidité ne nous étonne pas de la part de l'ancien ministre d'État, bien conscient que libre-échange et lutte contre le réchauffement climatique sont incompatibles. Fabien Gay l'a rappelé, il n'est pas besoin d'être un expert du GIEC pour faire ce constat : le fret mondial représente 10 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, et son volume devrait augmenter de 290 % d'ici à 2050. Le rapport neutre et dépassionné de la commission d'évaluation du CETA, remis au Premier ministre le 14 septembre 2017, l'a confirmé. Mais la France avait déjà décidé d'appliquer le CETA de manière anticipée dès le 21 septembre, sans attendre l'aval du Parlement. Une décision peu démocratique ! C'est à se demander d'ailleurs pourquoi le Gouvernement s'est donné la peine de commander un rapport le 3 juillet. Sans doute pour permettre à Nicolas Hulot de sauver la face en brandissant une recommandation du rapport visant à instaurer un veto climatique. Il va de soi que, sans rouvrir les négociations sur le CETA, l'entreprise s'annonçait juridiquement complexe. Il suffisait d'entendre les propos de votre collègue Brune Poirson, secrétaire d'État, pour s'en convaincre Nous avons sollicité la commissaire européenne au commerce, qui a indiqué être d'accord pour travailler sur le veto climatique ». Ce dernier prendrait « la forme d'une déclaration juridique interprétative, qui sera adossée à la partie consacrée aux investissements dans le CETA le confirmait dans cet hémicycle le 8 mars dernier : « Je ne vous le cache pas, nous devrons faire durant le printemps un véritable travail de conviction à la fois auprès de nos partenaires européens et évidemment de nos amis canadiens. »

nous pouvons voir que le monde ne s'est pas arrêté de tourner. Nous n'avons pas été envahis par un certain nombre de substances dont nous n'aurions pas voulu. S'agissant du veto climatique, la France a tenu la plume : nous avons transmis un projet de texte,

Si, sur le plan commercial, l'accord est présenté de façon positive, le moins qu'on puisse dire, c'est que, du point de vue environnemental - mon collègue vient de s'en faire l'écho - les inquiétudes persistent. Le calendrier de l'accord de Paris peut expliquer que ses conclusions ne se retrouvent pas dans le CETA, mais il est temps aujourd'hui qu'elles soient prises en compte. La France doit convaincre la Commission européenne de conclure un accord complémentaire prévoyant la neutralité du CETA en matière d'émissions de gaz à effet de serre, serre, l'interconnexion des marchés carbone, et une taxation spécifique sur le transport maritime. De même, nous attendons une déclaration interprétative précisant le sens à donner aux dispositions sanitaires et environnementales insuffisamment claires dans le traité, ainsi que l'application du principe de précaution. L'accord avec le Canada est un accord vivant. Il doit, avant que l'on nous propose de le ratifier, être amélioré. L'Europe doit exporter ses marchandises, mais aussi ses standards sociaux et environnementaux.

le plan d'action prévoyait que nous puissions compléter l'accord. Ce complément s'est concrétisé le 16 avril dernier, au moment où le Premier ministre Justin Trudeau est venu en France. Un partenariat avec neuf engagements très concrets a alors été signé. Par exemple, un travail commun est mené au sein de l'Organisation maritime internationale pour réduire les émissions du transport international.

très strictes, qui sont assorties d'un appareil de sanctions efficaces pouvant aller jusqu'à la révocation du juge par l'Union européenne et le Canada. Ces modalités devraient être adoptées courant 2019, dans tous les cas avant l'entrée en vigueur du tribunal d'investissement, laquelle

Le Canada n'est pas nécessairement le plus mauvais partenaire en matière environnementale. Cela dit, les inquiétudes persistent, en particulier sur la volonté d'adhésion de l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Nous aimerions savoir si la France a réussi à convaincre l'ensemble de ses partenaires pour avancer d'un même pas dans cette direction. Par ailleurs, pour ce qui concerne l'accord de règlement des différends, nous attendons un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne

Je pense au Brexit, au budget italien et aux tweets de M. Trump. Pour mon groupe, il est opportun de marquer notre attachement à un développement du commerce international régulé. Le groupe Union Centriste est favorable au CETA, raison pour laquelle nous souhaitons sa ratification par le Parlement.

» Ce n'est pas parce qu'on est favorable au développement du commerce qu'on ne souhaite pas une plus grande régulation. Nous préférons donc les termes « commerce régulé

avec, en toile de fond, pour l'agriculture canadienne, la possibilité d'exporter en Europe des denrées agricoles telles que la viande porcine et la viande bovine, alors que les conditions d'élevage sont radicalement différentes des nôtres.

cela fait un an jour pour jour que les produits canadiens entrent en Europe et en France, alors que l'accord n'a pas encore été ratifié par le Parlement. Monsieur le secrétaire d'État, comment pouvez-vous faire cela à nos agriculteurs et, surtout, aux consommateurs français ?

La cohérence, c'est de se dire que, dans cette mondialisation, nos filières agricoles ont beaucoup à gagner. Nous sommes en

le rappelle, pour la filière bovine, les contingents d'importation à droit nul concédés au Canada ont été fixés à plus de 45 000 tonnes, soit 0,6 % de la consommation européenne. le CETA prévoit que l'Union européenne puisse activer une « clause de sauvegarde », afin de réduire temporairement les quotas canadiens en cas de soudain « déséquilibre du marché d'un produit agricole ». Force est de le constater, la déstabilisation de la filière bovine risque de se révéler lente et progressive, dès lors que l'ouverture des contingents à droit nul ne sera complète qu'au bout de sept ans. Aussi la déstabilisation de la filière bovine ne devrait-elle pas, permettre l'activation de la clause de sauvegarde prévue par le CETA, celle-ci ne pouvant intervenir qu'en cas de déstabilisation soudaine et importante du marché. Néanmoins, lorsque ces quotas seront pleinement ouverts, nous avons de bonnes raisons de croire qu'ils deviendront véritablement attractifs pour la filière canadienne, qui se révélera dès lors structurellement plus compétitive que la filière française. En effet, si les contingents à droit nul devraient dans un premier temps rester limités et peu attractifs, de nombreux observateurs considèrent qu'une fois que les contingents de cette nature offerts au Canada auront atteint leur rythme de croisière, ils deviendront plus attrayants pour les exportateurs canadiens. donc deux questions à vous poser, monsieur le secrétaire d'État. Tout d'abord, que prévoit le Gouvernement pour accompagner les éleveurs une fois que tous les quotas seront totalement ouverts et que la filière canadienne sera complètement attractive

également porteur d'opportunités considérables, tant pour le boeuf que pour le porc. C'est la même chose pour l'accord qui a été conclu avec le Vietnam.

À ce stade, je pense utile de faire référence à la procédure d'équivalence, qui permettra aux Européens et aux Canadiens d'harmoniser certaines normes équivalentes, notamment en termes de protection de l'environnement.

dus à la pollution par les hydrocarbures, nous avions préconisé d'améliorer le fonctionnement du régime international d'indemnisation, en accélérant le traitement des demandes d'indemnisation en cas de sinistre de grande ampleur.

L'accord économique et commercial global, qui est entré en vigueur le 21 septembre 2017, permet la suppression progressive des barrières douanières entre l'Union européenne et le Canada, afin de faciliter l'accès des entreprises canadiennes et européennes aux marchés de la zone partenaire et de stimuler l'investissement des deux côtés de l'Atlantique. Ces échanges commerciaux sont particulièrement significatifs. Ils s'élèvent aujourd'hui à près de 60 milliards d'euros par an. À terme, l'accord pourrait permettre d'augmenter le volume global de ces échanges de 25 %, soit 12 milliards d'euros supplémentaires par an pour le PIB de l'Union européenne. En un an, la France a déjà bénéficié du CETA, avec une croissance de la valeur de ses exportations d'environ 5 %, notamment dans le secteur agroalimentaire ; par exemple, l'augmentation est de 8 % pour les fromages et produits laitiers et de 14 % pour les vins.

loin des fantasmes véhiculés par quelques adeptes du repli sur soi, le CETA ne modifie en rien les règles sanitaires propres à chaque État. Les verrous institutionnels appliqués aux mécanismes de coopération réglementaire permettront de préserver la souveraineté des deux partenaires, leurs modèles sociaux et leurs réglementations environnementales. Encore une fois, cet accord offre de véritables chances pour notre pays, notre économie et nos entreprises. C'est pourquoi je souhaite vivement que le Gouvernement lui apporte un soutien déterminé, à l'instar des douze États membres de l'Union européenne qui l'ont déjà ratifié. Je rentre tout juste du Canada,

nous ne sommes pas informés sur les conséquences d'une absence de ratification parlementaire. Qu'en est-il ? Où en est le Gouvernement dans son plan d'action aujourd'hui ? Une plus grande transparence et un effort d'information me semblent nécessaires.

européenne. Au mois de septembre, seulement 258 entreprises exportatrices françaises s'étaient enregistrées pour s'ouvrir sur le marché canadien, contre 410 en Belgique, 1 200 en Allemagne et 12 000 au Royaume-Uni

Une cinquantaine de réunions ont d'ores et déjà été organisées par les chambres de commerce sur les territoires. Il faut continuer et amplifier ce mouvement. Il me semble important de pouvoir

La séance est levée.